Madame la présidente,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

du scrutin. Par lettre en date du 10 avril 2018, le Gouvernement a demandé l'inscription à l'ordre du jour du jeudi 19 avril, le soir, et, éventuellement, du vendredi 20 avril, le matin et l'après-midi, de la suite de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Acte est donné de cette demande. L'ordre du jour appelle la désignation des vingt et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 L'ordre du jour appelle la désignation des vingt-sept membres de la mission d'information sur le développement de l'herboristerie et des plantes médicinales, des filières et métiers d'avenir, créée sur l'initiative du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen en application du droit de tirage prévu par l'article 6 du règlement. En application de l'article 8, alinéas 3 à 11, et de l'article 110 du règlement, la liste des candidats établie par les groupes a été publiée. Elle sera

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le mercredi 14 mars 2018, la commission mixte paritaire réunie sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, après deux lectures dans chaque assemblée, est parvenue à un accord. Je salue à ce titre la qualité du travail commun réalisé avec nos homologues de l'Assemblée nationale, en particulier avec le rapporteur du texte Sacha Houlié, de même que celui qui a été effectué avec le Gouvernement, dans un esprit très constructif. Trois dispositions étaient encore en discussion lors de cette commission mixte paritaire : la caducité de l'offre de contrat en cas de décès de son destinataire ; les clauses pouvant être contestées en raison d'un caractère prétendument abusif dans les contrats d'adhésion ; enfin, la révision judiciaire du contrat à la demande d'une seule des parties en cas de changement de circonstances imprévisible. La commission mixte paritaire a retenu la position du Sénat sur les deux premiers points et nous nous en sommes remis à celle de l'Assemblée nationale sur le troisième. La plupart des apports du Sénat en première lecture ont été conservés ; il est vrai que, pour ne pas contribuer à l'instabilité du droit, ils étaient limités à la correction des malfaçons et des difficultés d'interprétation les plus fortes. citons en particulier la nouvelle définition du contrat d'adhésion et le champ de la sanction des clauses abusives dans ces contrats ; la mise en cohérence de l'obligation précontractuelle d'information et de la définition de la réticence la meilleure articulation des règles en matière de capacité et de représentation avec le droit des sociétés ; les critères autorisant le paiement en devises sur le territoire français, en accord avec les pratiques jusque-là admises ; ou encore l'affirmation claire selon laquelle la loi nouvelle ne doit pas s'appliquer aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. La commission des lois avait par ailleurs levé plusieurs difficultés d'interprétation, sans modifier le texte, en précisant, dans le cadre des travaux préparatoires, le sens qu'il convenait de donner à certaines dispositions. Ces interprétations ont été partagées par le Gouvernement et l'Assemblée nationale. Sur la révision judiciaire du contrat pour imprévision à la demande d'une seule des parties, nous savons bien que cette innovation, critiquée, sera systématiquement écartée dans les contrats où les parties seront bien conseillées Cette innovation restera donc, à notre avis, sans grande portée. Ce débat aura eu le mérite de mettre en lumière le caractère éminemment politique de la réforme du droit des contrats, réalisée par par ordonnance au prétexte qu'elle était technique, alors qu'il s'agissait en réalité de faire de vrais choix politiques, dont le Parlement a été dessaisi et sur lesquels nous avons décidé de ne pas revenir. Cela nous donne matière à réflexion pour le futur, en particulier pour la réforme de la responsabilité civile, au moins aussi importante que celle du droit des contrats. Le Sénat s'en est d'ailleurs déjà saisi, puisque mon collègue Jacques Bigot et moi-même venons d'engager une mission d'information sur le sujet. La parole

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui au terme du processus de ratification de l'ordonnance réformant le droit des contrats, de la preuve et le régime général des obligations. C'est devant votre assemblée que s'était ouverte la phase parlementaire de cette procédure législative. C'est devant votre assemblée qu'elle s'achève aujourd'hui, traduisant le point d'aboutissement de cette réforme que

Mais au-delà de l'accord qui vous est aujourd'hui soumis, le succès de cette ratification tient, aux yeux des membres du Gouvernement, à la qualité des débats auxquels elle a donné lieu, ainsi qu'à l'esprit de responsabilité qui a animé les deux assemblées à chaque étape de la discussion. En effet, sans attendre la commission mixte paritaire, chacun a su faire un pas vers l'autre. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette tribune, mais je tiens à

Le texte qui vous est soumis est un texte exceptionnel à plusieurs égards. Il est d'une ampleur rare- près de 350 articles -et d'une technicité toute particulière, qui a conduit le rapporteur de votre commission des lois à mener un travail d'analyse tout à fait considérable. C'est surtout un texte fondamental pour les relations économiques, des plus usuelles aux plus exceptionnelles. Cet exercice de ratification présentait également un enjeu capital en termes de sécurité juridique. Il appartenait naturellement au Parlement de se saisir de l'ordonnance et d'en modifier les termes, s'il le jugeait nécessaire. Mais il fallait parallèlement prendre en considération le fait que ce nouveau droit des contrats était entré en vigueur depuis plus d'un an et que les praticiens se l'étaient d'ores et déjà approprié, au prix d'importants efforts d'adaptation compte tenu de l'ampleur que je relevais précédemment. Cet enjeu, monsieur le rapporteur, vous l'avez immédiatement saisi et ne l'avez jamais perdu de vue. Vous avez veillé à concentrer les débats sur les modifications qui vous sont apparues strictement nécessaires.

Les modifications apportées n'avaient, pour la grande majorité d'entre elles, qu'un seul objectif : préciser la loi pour renforcer la sécurité juridique. L'exigence de sécurité juridique a réellement guidé les travaux de votre commission des lois, qui a par ailleurs proposé de nombreuses lignes d'interprétation,

Au-delà de la correction de quelques malfaçons, les deux lectures ont permis aux deux assemblées de converger sur de nombreux points. Pour en donner quelques exemples, je pourrais citer la définition du contrat d'adhésion, figure contractuelle devenue incontournable, qui a fait son entrée dans le code civil et qui est désormais clarifiée le sort des sûretés en cas de cession de contrat ou de dette a, lui aussi, été précisé, tandis que le mécanisme de la réduction du prix a été rendu plus lisible.

de la disposition relative à la réticence dolosive, qui a été mise en cohérence avec la solution retenue en matière de devoir général d'information. Il en résulte que l'estimation de la valeur de la prestation est désormais exclue du champ de la réticence dolosive, afin d'inscrire dans la loi la jurisprudence.

Sur le premier point, le texte qui vous est aujourd'hui soumis définit clairement et opportunément le champ de la prohibition des clauses abusives. L'étendue de ce champ a donné lieu à un débat extrêmement soutenu. Au terme de vos travaux, celui-ci recouvre désormais les clauses non négociables au sein des contrats d'adhésion. Cette modification, qui ne remet pas en cause le caractère protecteur protecteur de cette disposition, est parfaitement cohérente avec les critères dégagés au cours de la navette sur la définition du contrat d'adhésion : c'est précisément la soustraction de ces clauses à la négociation qui justifie l'atteinte portée à la force obligatoire du contrat. Le second point majeur de débat porta sur les prérogatives du juge en matière d'imprévision. Le principe même de la révision du contrat pour imprévision n'a pas été remis en cause, démontrant ainsi le consensus existant sur l'utilité de cette innovation majeure de l'ordonnance pour adapter notre droit des contrats aux bouleversements économiques qui peuvent affecter leur exécution. Le seul point de désaccord résidait dans la faculté pour le juge de réviser le contrat à la demande d'une seule des parties. Le Gouvernement était et reste persuadé de l'utilité de prévoir cette option, sans laquelle l'efficacité du dispositif risquait d'être paralysée en cas de mauvaise foi de l'un des contractants. Les débats nourris sur ce sujet auront permis de rappeler, s'il en était besoin, le caractère supplétif de cette disposition et surtout d'en démontrer, au-delà de ces murs, l'utilité en certaines hypothèses, en ce sens que la rupture du contrat ne se révèle pas toujours la la solution économiquement la plus adaptée. Ainsi, au-delà de la confrontation des points de vue, nécessaire sur ces dispositions importantes, le dialogue constructif des chambres,

Votre assemblée s'en est d'ores et déjà saisie, puisqu'elle a confié à vos collègues François Pillet et Jacques Bigot une mission d'information sur ce projet, élaboré selon la même méthode ouverte et transparente que celui de la réforme des contrats. Je forme donc aujourd'hui le voeu que l'esprit de responsabilité et de compromis

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme nombre d'entre nous, je salue le compromis auquel la commission mixte paritaire est parvenue ; il va permettre de clore treize ans de réflexions. Si certaines réformes d'envergure nécessitent de s'inscrire dans le temps long, on peut raisonnablement considérer que celle-ci a souffert de certains temps morts législatifs et de son lot d'incertitudes ... Alors que nous nous préparons à ouvrir les discussions sur les chantiers de la justice, cette expérience devrait nous inviter à réfléchir à la question du recours aux ordonnances pour de telles modifications, qui sont de grande envergure et dépassent une simple codification à droit constant. Il est clair que le raccourcissement du mandat donné au Président de la République rend la conduite de tels chantiers plus délicate, dans des délais extrêmement courts, qui conduisent soit à négliger la consultation en amont, soit à léguer ces chantiers, inachevés, à la postérité. C'est une contrainte à laquelle Portalis a échappé Nous considérons que, dans ces conditions, le recours aux ordonnances ralentit le processus législatif global et expose inutilement les personnes tenues d'appliquer le droit au risque de revirements législatifs au moment d'une ratification intervenant après une alternance, surtout si l'ordonnance procède à des transformations substantielles. En ce qui concerne la ratification, toutefois, je crois que le succès de la commission mixte paritaire illustre le sens des responsabilités qui prévaut au Parlement, lorsqu'il s'agit de conduire des réformes de fond sans mettre en danger la sécurité juridique de nos concitoyens. En effet, le texte issu de la commission mixte paritaire répond aux objectifs fixés en 2016 par le précédent gouvernement au moment du dépôt de l'ordonnance : d'abord, le renforcement de l'accessibilité de notre droit des contrats, pour lutter contre l'éparpillement des normes que nous connaissions depuis 1804 ensuite, une plus grande protection de la partie la plus faible du contrat ; enfin, une modernisation de notre droit pour répondre à un souci d'attractivité économique. Cette dernière version permet un bon équilibre entre les différentes propositions de nos deux chambres,

À ce sujet, l'Assemblée nationale s'était montrée quelque peu réticente, invoquant notamment les contrats immobiliers, mais, selon nous, le maintien de la caducité garantit une plus grande clarté et sécurité juridique. C'est pourquoi nous nous félicitons du pas fait par l'Assemblée nationale en ce sens. que, après trois modifications, nous ayons trouvé un terrain d'entente sur les contrats d'adhésion. L'Assemblée nationale, qui, de prime abord, souhaitait étendre la possibilité d'utiliser le dispositif des clauses abusives à l'ensemble du texte, s'est également rangée à l'avis de notre chambre. La rédaction voulue par les députés aurait permis que toutes les clauses d'un contrat puissent être frappées de nullité, à l'exclusion de celles qui déterminent l'objet du contrat, comme le prix. Ils ont finalement accepté que cette disposition ne s'applique qu'aux clauses non négociables. Sur ce sujet, on peut considérer que la qualification en clause abusive ne dépend pas seulement du contenu de celle-ci. Elle s'apprécie surtout par rapport à l'équilibre général du contrat. Ainsi, un déséquilibre causé par une clause non négociable peut très bien être compensé par une clause négociable. Enfin, revenons sur l'article 8 : notre chambre était peu disposée à consacrer la théorie de l'imprévision dans notre droit civil. Je considère que cette disposition contribuera à apaiser les relations contractuelles, en permettant une demande de révision du contrat par l'une des parties en cas d'échec de la renégociation. Le recours Le recours au juge devrait également permettre de les pacifier : il faut voir cette mesure, non comme une contrainte, mais d'abord comme un appel aux parties à trouver un accord à l'amiable. Actuellement, la partie rencontrant des difficultés à exercer le contrat ne peut en demander la révision. Elle est même poussée à aller jusqu'au bout de celui-ci, quand bien même l'exécution du contrat est excessivement difficile pour elle et sa réalisation vitale pour son activité. elle ne peut pas y mettre un terme pour contracter avec un autre partenaire à un moindre coût. Faire en sorte, comme le souhaitait la Haute Assemblée, que les deux parties soient d'accord pour demander la révision aurait bloqué toute renégociation, la partie favorisée n'y ayant généralement aucun intérêt. La version La version proposée par les députés et intégrée dans le texte me paraît donc plus adaptée. Les membres du groupe du RDSE voteront donc ce texte, qui constitue un équilibre très acceptable et préserve la sécurité juridique de nos concitoyens. La

un triple objectif : la codification de la jurisprudence, qui s'était développée depuis deux siècles ; l'amélioration de la lisibilité, donc de l'accessibilité du droit des contrats ; enfin, le renforcement de l'attractivité du droit français vis-à-vis des entreprises, en clarifiant et en adaptant ce dernier aux enjeux de l'économie mondialisée. Je tiens ici à saluer sincèrement le travail colossal effectué par notre rapporteur François Pillet, ainsi que l'esprit de responsabilité qui a présidé à nos travaux, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, lors des deux lectures. Grâce à ce dialogue des chambres, marqué par la volonté de tendre vers le compromis, nous parvenons à un texte amélioré, dont l'équilibre et l'essence demeurent fidèles à ce que le Gouvernement souhaitait lui conférer.

la position du Sénat a été retenue, puisque le rapporteur de l'Assemblée nationale, Sacha Houlié, a notamment accepté de limiter l'application du dispositif des clauses abusives aux seules clauses non négociables. Sur le troisième point- la révision

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme je l'ai déjà dit lors des précédentes discussions générales, ce texte a deux mérites essentiels : premièrement, rendre le droit des obligations plus visible et plus accessible en y intégrant une foisonnante jurisprudence ; deuxièmement, renforcer la protection de la partie faible, en introduisant la notion de bonne foi à toutes les étapes de la conclusion du contrat et celle de vice du consentement pour tenir compte de la violence de la vie économique, qui- -ne fait pas de cadeau. Le texte permet ainsi de corriger les éventuels déséquilibres entre les parties et consacre le devoir général d'information. À l'issue de la commission mixte paritaire restaient trois points de discussion. restaient trois points de discussion. S'agissant de la caducité de l'offre de contrat en cas de décès de son destinataire, l'Assemblée nationale a suivi la version du Sénat, qui étend la caducité de l'offre en cas de décès de l'auteur ou du destinataire. Cette solution nous convient. S'agissant de la révision judiciaire du contrat en cas de changement de circonstances imprévisible, en revanche, c'est la version de l'Assemblée nationale qui a prévalu, version prévoyant une possible révision à la demande d'une seule des parties. Ayant soutenu cette position lors de nos discussions et défendu alors l'amendement déposé par Mme la garde des sceaux, je ne puis que me féliciter de ce choix, qui est conforme à l'esprit général des propositions de notre commission des lois, lois, visant, je le répète, à renforcer la protection de la partie faible. Le troisième point concernait la définition des clauses abusives dans un contrat d'adhésion. L'Assemblée nationale a accepté la version du Sénat, qui prévoyait de limiter l'application du dispositif des clauses abusives des contrats d'adhésion aux seules clauses non négociables, et non à toutes les clauses, comme le souhaitait l'Assemblée nationale au nom de l'intérêt des parties les plus faibles. En l'occurrence, je ne puis que regretter ce choix qui, encore une fois et sur ce point précis, est en contradiction avec l'esprit général dans lequel la commission des lois du Sénat a abordé la problématique contractuelle.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à la différence des pays placés sous le régime de la, la France est un pays de droit écrit au sein duquel sont garanties l'accessibilité de la norme et la sécurité juridique. paradoxalement, notre droit des contrats et notre régime des obligations souffrent, depuis de nombreuses années, d'une imprévisibilité et d'un manque crucial de lisibilité, plusieurs dispositions étant clairement obsolètes. civil, un projet de réforme du droit des contrats avait été annoncé. C'est ce long processus que nous allons aujourd'hui clore, en ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Sur la forme, et c'est aussi un véritable problème de fond, le Sénat s'était opposé de nouveau -et à juste titre !-au recours aux ordonnances, estimant que cette voie n'était pas justifiée pour une réforme qui n'était pas uniquement technique, mais reflétait aussi des choix de nature éminemment la marge de manoeuvre des parlementaires était d'autant plus réduite que nous avons dû ratifier cette ordonnance plus d'un an après son entrée en vigueur. En dépit de ces problèmes récurrents, le Sénat a fait preuve de responsabilité en s'attachant à clarifier le texte de l'ordonnance sans en modifier le sens, ni l'esprit. Sur le fond du sujet, nos deux assemblées se sont accordées sur le caractère essentiel d'une réforme unanimement saluée par les acteurs du droit. Cette ordonnance présente un double objectif il s'agit de renforcer, d'une part, l'attractivité du droit français, d'autre part, la sécurité juridique du droit des contrats, en améliorant tant sa lisibilité que son accessibilité. Le texte de l'ordonnance porte ainsi la consécration de mécanismes juridiques issus de la pratique, comme la cession de dettes ou la cession de contrats, tout en les simplifiant. Nos deux assemblées ont convergé sur de très nombreux points, en s'accordant sur la clarification de la définition du contrat d'adhésion et sur l'amélioration de la lisibilité du mécanisme de la réduction du prix. Les solutions innovantes introduites par l'ordonnance ont été évidemment les points les plus débattus. Deux d'entre elles, la prohibition des clauses abusives dans un contrat d'adhésion et la révision judiciaire pour imprévision, restaient encore en discussion lors de la commission mixte paritaire. Il s'agissait également de trouver un accord concernant la caducité de l'offre à la suite du décès de son destinataire. Sur ces trois sujets, la commission mixte paritaire est parvenue à la conclusion d'un accord, ce dont nous nous félicitons sincèrement. Je tiens ici à saluer particulièrement le travail accompli par notre rapporteur, François Pillet. de la caducité de l'offre de contrat en cas de décès de son destinataire, la position du Sénat a été suivie. Le silence de la loi sur ce sujet constituait une source d'incertitude pour les héritiers qui, après le décès d'un proche et en cas de litige avec l'auteur du contrat, devaient s'en remettre aux tribunaux.

Les dispositions ayant trait à la révision judiciaire du contrat pour imprévision ont suscité plus de débats. Il était question de savoir si le pouvoir de révision pouvait émaner d'une des deux parties uniquement, ce qui, pour le Sénat, constituait un gage d'insécurité juridique. Toutefois, dans la mesure où cette hypothèse devrait heureusement rester théorique, sinon lettre morte, il a été décidé de se rallier à la position de l'Assemblée nationale, dans un esprit de compromis auquel nous nous sommes pleinement associés. Mes chers collègues, aujourd'hui, je serai brève, soulignant que le projet de loi ratifiant cette ordonnance offre à nos partenaires économiques un cadre sécurisant et dote la France d'instruments juridiques modernes et lisibles.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, l'ordonnance du 10 février 2016 a procédé à une refonte de grande ampleur du code civil. Cette réforme, qui concerne le droit des contrats, le régime général des obligations et le régime de la preuve des obligations, était très attendue. Renforcer la sécurité juridique et l'attractivité du droit des contrats, le moderniser, le rendre plus lisible sans le bouleverser, l'adapter aux enjeux contemporains en considérant l'exigence d'efficacité économique et en consolidant la jurisprudence, tels sont, en effet, les objectifs de cette réforme nécessaire. Le 14 mars dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord. Trois dispositions étaient encore en discussion : la première, sur la caducité de l'offre de contrat en cas de décès de son destinataire la deuxième, sur les clauses pouvant être contestées en raison d'un caractère prétendument abusif dans les contrats d'adhésion ; la troisième, enfin, sur la révision judiciaire du contrat à la demande d'une seule des parties en cas de changement de circonstances imprévisible. La commission mixte paritaire a retenu la position du Sénat sur les deux premiers points et celle de l'Assemblée nationale sur le troisième. Je souhaite remercier ici, à cette tribune, le rapporteur de ce texte, très technique

civil, Jean-Étienne-Marie Portalis, dont la statue domine cet hémicycle, disait : « Les lois ne sont pas de purs actes de puissance. Ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois, qu'elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites Oui, notre code civil doit pouvoir refléter l'état réel du droit positif, qui a évolué sous l'oeuvre de la jurisprudence et de la doctrine depuis 1804. Notre groupe votera donc en faveur de la ratification de l'ordonnance du 10 février 2016

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette réforme de grande ampleur du code civil concernant le droit des contrats, le régime général des obligations et le régime de la preuve des obligations apparaît bien nécessaire, tant ce domaine a évolué depuis 1804, sous l'oeuvre de la jurisprudence et de la doctrine Le 14 mars dernier, la commission mixte paritaire a procédé à l'examen des dispositions restant en discussion concernant trois articles. À l'article 4, le Sénat a souhaité établir la caducité de l'offre en cas de décès du destinataire. La commission mixte paritaire a retenu sa position. À l'article 7, le Sénat entendait limiter l'application du dispositif des clauses abusives des contrats d'adhésion aux seules clauses non négociables. L'Assemblée nationale avait une position différente : elle souhaitait étendre cette possibilité, dans l'intérêt des parties les plus faibles, à toutes les clauses du contrat. Mais dès lors qu'un accord avait été trouvé sur l'ensemble contractuel défini à l'article 2, l'Assemblée nationale a rejoint le Sénat sur cet article 7. Une difficulté demeurait toutefois sur l'article 8, qui modifie l'article 1195 du code civil et traite du régime de l'imprévision. Le Sénat prévoyait de donner pouvoir de révision du contrat au juge à la demande des deux parties, alors que l'Assemblée nationale souhaitait que la demande puisse émaner de l'une des deux parties seulement. Le Sénat jugeait cette faculté contraire à la sécurité juridique. Je voudrais saluer, à cette tribune, la qualité des travaux de notre rapporteur, François Pillet, comme son pragmatisme sur cette question. Ainsi, je me réjouis qu'il ait accepté la rédaction de l'Assemblée nationale, considérant que cette disposition est supplétive et restera de l'ordre de l'hypothèse. Cette innovation sera donc sans grande portée. Avant de conclure, je voudrais rappeler qu'en 2015 le Sénat tout entier s'était opposé à ce que le Gouvernement procédât par ordonnance à la réforme la plus ambitieuse du code civil depuis 1804. Il apparaît donc inconcevable que, pour la future réforme du droit de la responsabilité civile, le Gouvernement utilise la même méthode ! Madame la ministre, mes chers collègues, cette réforme du droit des contrats répond à deux nécessités : la codification de la jurisprudence qui s'est développée depuis deux siècles et l'adaptation

la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'élection des représentants au Parlement européen Dans la discussion du texte de la commission, nous sommes parvenus à l'amendement n° 70 rectifié, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme le soulignaient certains de nos collègues du groupe Les Républicains dès l'examen de notre proposition de loi visant à rétablir la circonscription unique pour les élections européennes, la désaffection de nos concitoyens pour ce scrutin comporte également des « causes exogènes », non liées à la nature du scrutin. La difficulté pour s'informer de l'actualité politique européenne en est une, dès lors que la plupart des médias « généralistes », à l'exception d'Arte, se concentrent sur le suivi de la vie politique nationale. Certains sites Certains sites internet d'actualité très bien documentés existent également, mais ils n'attirent pas des publics très nombreux. Nous qui sommes régulièrement chargés de la transposition des directives et de la mise en conformité de notre droit aux règlements adoptés au niveau européen, nous sommes conscients de l'impact du travail réalisé en amont par le Conseil et le Parlement européens sur le droit s'imposant aux Français, par exemple, tout récemment, en matière de protection des données personnelles. Dans de nombreuses matières, il serait utile de déplacer le débat public au moment des négociations au sein de l'Union européenne, et non plus au stade de la transposition, moment où les capacités d'amendement de l'Assemblée nationale et du Sénat sont considérablement réduites. Cette anticipation permettrait une expression de la pluralité des opinions françaises au sein du Parlement européen, là où, au Conseil, le Gouvernement continuerait de représenter sa position. Or de tels débats ne peuvent intervenir sans une information régulière et continue sur l'actualité législative européenne, susceptible de faire réagir nos concitoyens. Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons cet amendement, qui vise à inscrire dans les cahiers des charges des grands médias publics des dispositions pour la promotion de l'information relative à l'actualité politique européenne, en plus de celles qui sont liées à leur mission éducative, ou encore de celles qui sont relatives à la lutte contre la discrimination et à la lutte contre le dopage, comme la loi de 1986 le prévoit également.

Claudine Kauffmann. Au moment où d'importants sacrifices sont demandés à nos concitoyens pour équilibrer les comptes publics, il convient de donner l'exemple en réduisant les dépenses électorales et, corrélativement, les remboursements à la charge de l'État. De plus, l'abaissement du plafond des dépenses permet de réduire les séquelles des distorsions démocratiques qui existent entre les listes selon les moyens financiers dont elles disposent.

qui correspond au plafond actuel non majoré- 1 150 000 euros -multiplié par le nombre de circonscriptions- huit. Une analyse des comptes de campagne permet de constater une baisse de 19 % des dépenses globales déclarées par les candidats en 2009 en 2014. La liste la plus dépensière en 2009 a engagé environ 900 000 euros pour sa campagne. En 2014, ce montant était de 700 000 euros. Il existe donc une dynamique à la modération des dépenses électorales qui constituent de l'argent public au travers de la défiscalisation des dons et du remboursement forfaitaire versé aux listes obtenant 3 % ou plus des suffrages exprimés. Au-delà de la baisse de 10 % de ce plafond en raison de l'abrogation de la majoration, la nationalisation du scrutin par une liste unique va induire mathématiquement d'importantes économies d'échelle. J'ai lu, dans le rapport de la commission, que cette proposition de modération des dépenses électorales serait sans effet réel. Or la nationalisation du scrutin va entraîner une mainmise des formations politiques, dont les trésoriers vont faire un calcul simple 9 200 000 euros de plafond multipliés par le taux de remboursement de 47,5 %, soit un montant de près de 4,4 millions d'euros sur lequel ils vont baser l'emprunt de leur liste Il est donc proposé de fixer ce plafond à 7 200 000 euros, soit 900 000 euros multipliés par l'ancien nombre de circonscriptions- huit. À plus d'un an du scrutin, cette diminution n'est pas de nature à porter atteinte à l'exercice du droit de suffrage garanti par l'article 3 de la Constitution.

Je tiens simplement à préciser que le Gouvernement a prévu dans ce texte des dispositions spéciales pour faciliter la campagne électorale des candidats d'outre-mer. Ainsi, le plafond des dépenses est augmenté de 2 %, soit 184 000 euros supplémentaires, pour prendre en compte les frais de déplacement et de transport depuis les outre-mer.

dans le projet de loi par le Gouvernement. Tous ceux qui se sont occupés, une fois ou l'autre, du financement d'une campagne électorale comprendront de quoi je parle. Aujourd'hui, un parti politique peut contribuer aux dépenses d'une campagne électorale.

se sont abstenus en France. Ce fait est très alarmant. En effet, par sa nature même, le projet européen convoque les générations futures, puisqu'il se définit comme un mouvement progressiste vers la construction d'institutions stables destinées à assurer une paix pérenne en Europe. La jeunesse est également au coeur du projet Erasmus, qui a commencé en 1987 et qui est destiné à permettre des échanges universitaires et à promouvoir les rencontres entre jeunes Européens. Cette abstention condamne notre jeunesse à un cercle vicieux moins elle prendra part aux élections européennes, moins elle permettra de dessiner une Europe conforme à ses aspirations ; or moins l'Europe se conformera à ses aspirations, moins la jeunesse votera aux élections européennes. Face à ce phénomène, il convient de prendre des mesures particulièrement fortes pour inciter nos concitoyens, en particulier les jeunes,

ou même celle des formalités du vote par procuration, compte parmi les facteurs qui les dissuadent de voter. C'est pourquoi nous proposons de leur ouvrir le droit de vote à distance, et même de manière électronique, lorsqu'ils poursuivent leurs études dans un département différent de celui de leurs parents. Il ne s'agit en réalité que du point de départ d'une longue réflexion,

madame la ministre, n'est offerte qu'aux Français établis hors de France, du fait de leur éloignement, et cela seulement pour les élections dans des circonscriptions comprenant uniquement des électeurs

Grand. Selon le même principe de la représentation territoriale minimale, nous proposons d'interdire qu'une région soit surreprésentée sur une liste de candidats en imposant qu'aucune région ne puisse fournir plus d'un cinquième des candidats

mais j'estime que garantir la présence d'un représentant de chaque région est une manière de responsabiliser les élus devant leur électorat.

plutôt que de les pousser à diluer leur vote dans les circonscriptions d'autres pays.

y compris à ceux qui ont été retirés, ce qui fait gagner du temps à tout le monde ! Aux termes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le suffrage est libre.

des candidats à une région française, alors que c'est une liberté. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les modalités proposées, la commission a considéré qu'il y a contradiction entre l'objet même du projet de loi, qui a été approuvé avec l'article 1, et tout système qui contraindrait la composition des listes.

on pourrait constater que certaines régions, démographiquement, pèsent trois ou quatre fois plus lourd que d'autres ; par conséquent, instaurer une égalité de représentation entre ces régions, au défi de la réalité démographique, ce serait également

n° 19 rectifié, d'imposer que les treize régions métropolitaines et les outre-mer aient tous un représentant dans le premier cinquième de la liste,

c'est se priver d'une liberté et d'une capacité réelle d'équilibre bien choisi au sein d'une liste. Par ailleurs, comme le code électoral n'impose comme critère d'éligibilité, outre la majorité et la capacité juridique, que la qualité d'électeur, sans considération de la commune d'inscription ou de résidence, je puis vous confirmer, mesdames, messieurs les sénateurs, que au regard du principe de liberté des candidatures. Je ne doute pas, comme je l'ai dit hier, que les différentes listes disposeront de candidats représentant la diversité des territoires, au même titre qu'elles présenteront des candidats aux profils variés, qui représenteront même, peut-être, des courants différents au sein même d'une famille politique- cela peut arriver En outre, je rappelle que les représentants français au Parlement européen ont vocation à y représenter, non pas notre diversité territoriale,

durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ce même droit est ouvert au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé de l'outre-mer, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. L'article 9 prévoyait quant à lui que les déclarations de candidature résultaient du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'État. Dès lors que l'ensemble des déclarations résultera désormais d'un dépôt au ministère de l'intérieur, il est proposé, par cohérence, de supprimer la faculté laissée au ministre chargé de l'outre-mer de contester l'élection. En effet, le ministère de l'intérieur assure sur tout le territoire le maintien et la cohésion des institutions du pays. Il a notamment pour mission d'élaborer et de faire respecter les règles garantissant aux citoyens l'exercice des libertés publiques, notamment par le suffrage universel. Dans ces conditions, le

Ainsi, pour les élections européennes, l'article 9 de loi du 7 juillet 1977 prévoit que, à la suite de sa signature, « chaque candidat appose la mention manuscrite suivante La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) L'article 14 de cette même loi précise les modalités du retrait des listes complètes avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature. Cette déclaration de retrait doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste. Afin de sécuriser les retraits comme les dépôts de candidature, il est proposé de prévoir l'apposition d'une mention manuscrite manifestant expressément l'accord du candidat pour le retrait de la liste. La signature ne suffit pas. Quel est l'avis de la commission

88-1 du code électoral punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi. Il est proposé d'appliquer une sanction similaire à tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui se serait porté candidat sur une liste sur la base de déclarations frauduleuses- fausse adresse, faux nom, candidature simultanée dans un autre État membre, inéligibilité dans son pays Il ne s'agit pas là de la sanction pour inscription pour fraude sur une liste électorale.

L'article 24 de la loi du 7 juillet 1977 fixe les modalités de remplacement des députés européens, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Afin de respecter la parité, il est proposé de prévoir un remplacement par le candidat de même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu, conformément à l'ordre de cette liste. Il s'agit là d'une disposition déjà applicable pour l'élection des conseillers communautaires.

lorsqu'un siège devient vacant, c'est le premier candidat non élu de la liste qui vient en succession, quel que soit son sexe.

L'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 définit les missions des sociétés nationales de programme qui composent le secteur public de la communication audiovisuelle : France Télévisions, Radio France et les chaînes en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Il prévoit notamment que celles-ci « favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté », mais aussi d'autres missions plus spécifiques encore, comme la promotion de langues régionales ou le développement de la création artistique. Selon l'esprit qui nous anime depuis le début de l'examen de ce projet de loi, il nous a semblé nécessaire d'inscrire la dimension européenne du débat démocratique et de la citoyenneté dans cet article, afin d'inciter ces médias à familiariser davantage les citoyens aux enjeux européens, notamment à l'actualité législative européenne. Il existe un véritable besoin d'information de nos concitoyens, pour qui le fonctionnement des institutions européennes reste assez opaque. Au vu des programmes actuellement proposés par les chaînes publiques, la dimension européenne du débat démocratique ne va pas de soi, malgré le renforcement des prérogatives attachées à la citoyenneté européenne. Cet amendement vise également à ne pas cantonner les débats relatifs à l'Union européenne aux seules périodes de campagnes électorales, ce qui contribue, selon nous, à des positions électorales pro ou anti-européennes. Un tel travail de fond d'analyse et d'information devrait permettre à terme de distinguer, dans l'esprit de nos concitoyens, l'outil- les institutions européennes -et le fond- les programmes politiques qui sont mis en oeuvre par le biais de cet outil. Il est en effet urgent de transférer le débat idéologique de l'existence de ces institutions vers les politiques qu'elles permettent de mettre en oeuvre.

? Madame la sénatrice, le Gouvernement partage pleinement l'ambition de renforcer le caractère européen du scrutin. C'est précisément ce qui l'a conduit à réformer la circonscription d'élection des représentants au Parlement C'est également parce qu'il a conscience de la nécessité de consolider le dispositif de campagne officielle au regard des impératifs d'équité et de représentativité

par la loi de 1986 celles de favoriser le débat démocratique dans les institutions européennes excède non seulement le cadre du présent texte, mais aussi son principal objet, le Parlement européen, car ces obligations seraient applicables même hors campagne électorale. En outre, il n'est pas évident de déterminer précisément ce que recouvre la notion de débat démocratique dans les autres institutions de l'Union que

Bien qu'il ne s'agisse pas de l'un des objectifs explicites de ce projet de loi et que les retombées ne se manifesteront vraisemblablement pas dès 2019, il me paraît nécessaire de s'attaquer à ce phénomène en modifiant les dispositions relatives à l'éducation morale et civique dans le code de l'éducation.

aux élections européennes des futures générations. Les ajouts que je propose ont, me semble-t-il, toute leur place au sein de la définition de l'éducation morale et civique actuelle.

l'article 7 du projet de loi prévoyait que, indépendamment des négociations européennes conduites en vue de créer une circonscription européenne unique au sein de laquelle des représentants seraient élus sur des listes transnationales, la présente loi entrerait en vigueur lors du prochain renouvellement des représentants français au Parlement européen. Cela signifiait que le texte entrerait en vigueur à ce moment-là, sans que l'aboutissement, ou la poursuite des négociations en la matière ne modifie la portée et les dispositions du texte. Votre commission a malheureusement supprimé la mention relative aux listes transnationales, ce que le Gouvernement regrette. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet est essentiel pour la démocratie et pour l'Europe, puisqu'il vise à créer un lien direct entre les citoyens et l'Europe en leur permettant d'élire des représentants au Parlement européen qui, au-delà d'être français, allemands, suédois ou maltais, sont des représentants européens, élus sur les projets qu'ils portent pour l'Europe, selon leur sensibilité politique.

au sein duquel les citoyens de plusieurs pays se rejoindraient pour porter un projet politique commun et confronter leurs idées à celles d'autres citoyens de l'Europe défendant un projet différent.

Ce projet fait toujours l'objet de négociations entre les États membres. Si nous avons pris acte du vote du Parlement européen en février dernier, nous rappelons qu'il ne portait pas sur le projet de révision de l'acte électoral européen, dont nous avons beaucoup parlé hier, pour lequel la France a proposé la création de ces listes transnationales. Il ne signifie donc pas, pas plus que la suppression de cette mention à l'article 7, que ce projet ne verra pas le jour. Je rappelle que

C'est dans cette perspective que le Gouvernement continuera à défendre cette idée, pour ne pas dire cet idéal, aussi bien en France qu'à l'échelon européen, afin qu'elle traduise de manière concrète

fondamental par ailleurs. Il s'agit d'un symbole permettant à ceux qui sont motivés par la construction d'un projet européen, rassemblant l'ensemble des citoyens de l'Union, de l'élaborer et de le porter dans de meilleures conditions.

La rédaction initiale de l'article 7 s'inscrivait dans la logique développée par le Président de la République, lequel souhaite faire évoluer l'Union européenne vers une structure fédérale au sein de laquelle les États-nations seraient marginalisés.

l'ai rappelé au début de notre discussion, chaque État légifère sur les modalités de l'élection de ses représentants au Parlement européen, à l'intérieur d'un cadre fixé par un acte européen, dont je rappelle d'un mot la genèse.

nécessaire. Or il n'y a pas de proposition sur la table, puisque la procédure d'adoption d'un nouvel acte européen n'est pas commencée. Le chef de l'État a pris des contacts, il a lancé des propositions.

Une majorité de sénateurs du groupe Les Républicains a soutenu une autre approche, l'ancrage régional, qui n'est pas la panacée, mais qui serait dans tous les cas un moindre mal pour essayer de renforcer le lien entre les citoyens et l'Europe. les grands pays, sauf l'Espagne, ont une circonscription régionale. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Italie et de la Pologne. Pologne. Songeons que l'Occitanie a la taille de l'Irlande et la Nouvelle Aquitaine celle de l'Autriche, que la France est un pays de 65 millions d'habitants qui élira au moins 74 députés, voire plus, et que nous prenons le risque d'élire des députés hors sol. Nous avons aussi beaucoup parlé, pendant ces débats, de la France ultramarine. La situation de la France ultramarine a été bien expliquée par notre collègue Michel Magras et par nos autres collègues ultramarins. Si nous n'avons pas voté les amendements visant à créer une circonscription ultramarine, c'est qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une circonscription unique, qui créait un système binaire ne pouvant pas nous satisfaire. L'amendement que j'ai présenté visait à créer une circonscription ultramarine et douze circonscriptions pour la France métropolitaine. Nous nous réjouissons malgré tout de l'adoption de l'amendement n° 30 rectifié, qui permettra d'intégrer les parlementaires européens dans le calcul du temps d'antenne de la campagne officielle. Je regrette, pour conclure, l'absence d'ancrage régional. Certes, le débat fut noble. Nous avons parlé de notre projet sur l'Europe, de notre volonté d'Europe. Nous avons parfois mélangé, dans les débats, carottes et navets, mais nous sommes parvenus à un rapport noble,

entre citoyens, territoires et élus de la République. Ce qui vaut pour les sénateurs doit valoir aussi pour les députés européens.

regrets, ces espoirs déçus, nous constatons que le fait de revenir à une circonscription nationale permet aux différentes manières de voir l'avenir de l'Europe, l'avenir de la France en Europe, de s'incarner

je ne paraphraserai pas son propos, mais reviendrai sur un élément précis qui explique pourquoi je ne voterai pas ce texte. La modification d'un mode de scrutin n'est jamais anodine. Il y a parfois, souvent même, des arrière-pensées politiques. Je ne fais pas ce procès à Mme la ministre dans le cas présent. À M. Macron ! Néanmoins, ces dernières années,

et force est de constater que cela n'a pas eu un effet positif sur l'abstention. Or j'ai bien entendu votre argument, madame la ministre : vous souhaitez, et c'est notre souhait à tous, que les citoyens reviennent vers les urnes.

pas électorale mais politique, c'est effectivement la réémergence d'un débat national sur l'Europe- je n'ai pas dit un débat nationaliste, c'est le droit des nationalistes de l'avoir. Il s'agit que l'on parle d'Europe à l'occasion des élections européennes.

le représentant centriste de l'époque, que j'estime beaucoup, s'est présenté quasiment comme un pré-candidat à l'élection présidentielle. La seule liste que j'ai eu la chance d'accompagner a parlé d'Europe et a fait un très bon score ! Déjà, ne détournons pas l'objet de l'élection. Que l'on soit pour

pour explication de vote. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les circonscriptions interrégionales n'ont pas permis de renforcer la proximité des électeurs avec leurs élus. Nombreux sont les citoyens, pour ne pas dire la très grande majorité, qui ignorent encore le nom de leurs représentants au Parlement européen. De plus, la participation n'a pas augmenté depuis la réforme introduite en 2003. Le découpage actuel n'a pas de cohérence au regard de la nouvelle carte des régions sur le territoire hexagonal instituée par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Un découpage n'ayant plus aucun lien avec le découpage administratif existant est de nature à complexifier la compréhension d'un scrutin déjà peu apprécié des électeurs. Enfin, le choix d'un scrutin à circonscriptions multiples éloignerait la France du modèle majoritaire dans l'Union européenne, celui d'une circonscription nationale unique adopté par vingt-deux des vingt-sept États membres.

Il souhaitait conserver un lien de proximité entre les électeurs et les élus. La grande majorité de notre groupe est donc favorable au projet de loi, qui vise à rendre le scrutin plus visible et permet la pédagogie pour favoriser l'image de l'Europe et convaincre les Français afin que l'Europe soit un projet d'avenir partagé. La parole

unique ait été rétablie comme cadre de l'élection des représentants de nos concitoyens au Parlement européen. J'ai eu l'occasion de développer les raisons pour lesquelles nous étions favorables à cette mesure.

ne nous invitent pas à voter en sa faveur. Le premier, c'est le maintien du seuil de 5 % pour accéder à la répartition des sièges, que seuls neuf pays européens ont adopté,

officielle, ce qui va, je le répète, favoriser les partis dominants et renforcer notamment l'influence des médias et des instituts de sondage. À l'inverse,

explication de vote. Le groupe Union Centriste se réjouit de la probable adoption de la liste nationale, si, dans quelques instants, nous sommes cohérents avec les votes que nous avons exprimés sur les articles. Notre bonheur serait encore plus complet si la voix de nos collègues d'outre-mer avait été entendue, ce qui nous conduira à exprimer, en leur nom, un vote négatif pour la question de la spécificité ultramarine. Sur le fond, qui est la manière dont notre pays aborde son rôle en Europe, nous aurions surtout souhaité que les listes puissent être transnationales ou transeuropéennes. Nous savons bien que ce n'est pas possible en l'état des équilibres politiques au sein du Parlement européen, puisque nous sommes dans un domaine qui relève de la codécision. Nous considérons en tout cas avec réalisme que la liste nationale

D'ailleurs, c'est un peu un rendez-vous de l'Histoire : depuis que l'Europe existe, c'est la première fois que cette élection va se passer dans un contexte politique européen complètement différent. Le Brexit Le Brexit nous oblige à apporter d'autres réponses à nos populations, aux acteurs économiques. L'ambition européenne que nous devons afficher et, surtout, faire partager à nos concitoyens

Je voudrais redire ici qu'il y a deux politiques essentielles au niveau de l'Union européenne : la politique agricole commune et la politique de cohésion des territoires.

et des parlementaires sortants, laissant penser que le débat ne se jouait pas au niveau des questions d'ordre géographique. Voilà qui est, me semble-t-il, tout à fait symptomatique de l'esprit qui anime ce texte

Pour l'avenir, le texte ne changera rien, il est purement cosmétique. Il ne servira qu'à une chose : donner un peu plus de liberté aux partis politiques pour maîtriser l'offre politique. Très bien ! Et tout cela au détriment de l'expression véritable du suffrage universel. Je me permets de vous annoncer, sans prendre trop de risques, le fiasco du 26 mai 2019. J'imagine déjà, sur les plateaux médiatiques- et sur internet ! -, les pleureuses dénoncer, avec beaucoup d'hypocrisie, la faiblesse de la participation électorale.

il aurait été anormal, à l'occasion de ce vote, que la principale victime n'eût pas fait entendre sa voix. Si la circonscription unique a existé, plusieurs circonscriptions ont été ensuite instaurées : « progrès », disions-nous à l'époque. L'Union européenne a même jugé bon de créer ce qu'on a appelé les PTOM, les pays et territoires

puisque ces mêmes zones ultrapériphériques n'ont aucune chance de se voir représentées. J'en prends bonne note. Les Ultramarins de mon groupe voteront contre ce texte, en toute cohérence ont tenus dans ce débat. Bravo ! Je suis très amer. Nous reviendrons un jour, je vous le promets. Ce n'est qu'une péripétie, certes grave, mais tout ce qui se fait peut être défait.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

que le prochain scrutin mobilisera davantage les citoyens. Je suis sûre que toutes les forces politiques ici présentes mettront un point d'honneur à porter haut les enjeux européens, dans le cadre de la future campagne. Voici